La séance est reprise. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour un rappel au règlement. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, demain, le Parlement sera saisi d'une déclaration du Gouvernement sur la mise en place de l'application StopCovid suivie d'un vote dans chaque assemblée en vertu de l'article 50-1 de la Constitution. Comment ne pas être surpris de la réapparition de ce petit serpent de mer, alors que beaucoup tenaient ce projet pour enterré, car trop tardif, inutile et efficace ? Comment, surtout, ne pas s'élever contre la place réservée au Parlement dans la mise en oeuvre de ce système numérique, qui soulève de lourds problèmes en matière de libertés publiques ? Il nous sera demandé de nous prononcer demain soir, alors que le Gouvernement a déjà annoncé que l'application était prête à être mise en oeuvre dès ce week-end. Certes, M. Cédric O conditionne cette mise en oeuvre au vote du Parlement, mais il exerce dans le même temps une pression difficilement acceptable en tentant de présenter le vote comme acquis et la mise en place de StopCovid comme évidente. Monsieur le président, nous l'avons déjà constaté après le vote négatif du Sénat sur le plan de déconfinement, les votes qui ne sont que de simples avis, à la différence du vote de confiance à l'Assemblée nationale,

Pourquoi donc annoncer avant même les débats la mise en oeuvre de StopCovid dès vendredi soir ? Pourquoi une telle obstination, une telle précipitation de dernière minute, alors que beaucoup estiment qu'elle n'a pas d'utilité ? La vérité est peut-être ailleurs Selon Cédric O, l'application « pourrait être disponible dans les magasins Apple et Android dès ce week-end ». Vraiment, le naturel de la « start-up nation » revient toujours au galop avant tout, le commerce toujours, avec la promotion, une fois de plus, des géants du numérique, alors qu'il s'agit d'une mission régalienne de protection de la santé publique

Sénat avait voté à la quasi-unanimité un amendement prévoyant, sur mon initiative, un taux de TVA réduit à 5,5 % sur les masques de protection, sur les gels hydroalcooliques et non hydroalcooliques de protection, ainsi que sur les équipements de protection.

est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne Notre séance se déroule dans les conditions de respect des règles sanitaires mises en place depuis le mois de mars. Je rappelle que l'hémicycle fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection avant et après chaque séance. Il en est de même pour les micros après chaque intervention. J'invite chacune et chacun à veiller au respect des distances de sécurité. Les entrées et les sorties de la salle des séances, pour les sénateurs, devront exclusivement s'effectuer par les portes situées au pourtour de l'hémicycle. Je rappelle également que tous les orateurs, y compris le Gouvernement, s'exprimeront depuis leur place, sans monter à la tribune.

mesdames, messieurs les sénateurs, voilà maintenant un peu plus de deux semaines que la France sort progressivement du confinement. Pendant longtemps, nos concitoyens ont attendu avec inquiétude ou espoir, parfois même les deux, la date fatidique du 11 mai. Ils sont désormais dans l'attente des futures étapes de ce déconfinement. Nombreux sont ceux qui veulent savoir si les restrictions apportées à la liberté de circulation seront levées ou allégées, si les bars, les cafés, les restaurants rouvriront leurs portes et s'ils pourront partir en vacances cet été. Retrouver ce qui fait au fond le sel de la vie sociale, reprendre une vie plus normale, tel est aujourd'hui le souhait de nos concitoyens. Nous devons nous réjouir de ces impatiences qui manifestent un puissant désir de retrouver le vivre ensemble. Dans le même temps, nous ne pouvons pas ignorer que cette période est source de contraintes, voire d'angoisses. Il est vrai que, pour un certain nombre de nos concitoyens, le confinement a pu paraître protecteur à bien des égards : d'un point de vue économique, puisqu'un salarié sur deux a été placé en chômage partiel ; d'un point de vue social, puisque d'importants filets de sécurité ont été mis en place pour accompagner les plus fragiles ; et d'un point de vue sanitaire enfin, puisque chacun était appelé à rester chez soi, loin du virus. Au désir de se retrouver répond donc l'inquiétude du jour d'après. Y aura-t-il une seconde vague ? Les entreprises seront-elles suffisamment résilientes ? Les emplois seront-ils préservés ? La sécurité de tous sera-t-elle toujours assurée ? Face à ce paradoxe auquel chacun d'entre nous est confronté, nous devons avancer sur une ligne de crête, ajuster les dispositifs et faire preuve d'agilité. Souvenons-nous que se précipiter signifie étymologiquement tomber la tête en avant. Faisons preuve de prudence, c'est ce que souhaite le Gouvernement, et de pragmatisme. Telle est la philosophie de ce projet de loi. Il vise à répondre à une multitude de questions et d'impératifs, ce qui explique son caractère singulièrement protéiforme. Il s'agit tout d'abord d'un projet de loi qui vise à garantir la continuité du service public. Tel est le sens des mesures tendant au maintien en service d'un certain nombre de militaires ou encore de l'augmentation du plafond de jours de mobilisation des réservistes de la police nationale. Je pourrais aussi citer la possibilité d'engagement de la réserve civique auprès des entreprises chargées d'une mission de service public. Ce projet de loi contient aussi des mesures destinées à permettre à l'administration de mener à bien des réformes que vous avez votées. Vous ne l'ignorez pas, l'administration a dû suspendre un certain nombre de ses activités en raison du confinement, parce qu'elle a notamment réorienté ses moyens vers la gestion de la crise sanitaire. Je pense ici au ministère des solidarités et de la santé. C'est la raison pour laquelle certaines réformes telles que celles du divorce, du versement des pensions alimentaires ou encore de la justice pénale des mineurs doivent être reportées pour être mises en oeuvre dans de bonnes conditions. Il en va de même pour certaines réformes intéressant Mayotte, la Martinique et la Guadeloupe, mais aussi la Polynésie française. Je sais que la ministre des outre-mer s'en est expliquée. Par ailleurs, ce projet de loi a pour objectif de faciliter la reprise de notre vie économique et sociale, tout en s'attachant à maintenir les droits des salariés. Tel est le sens des mesures visant à simplifier le recours au prêt de main-d'oeuvre ou encore la possibilité pour les travailleurs saisonniers de demeurer trois mois supplémentaires sur le sol national. La commission des affaires sociales a également adopté des amendements visant à limiter dans le temps les dispositifs dérogatoires tendant à assouplir les règles relatives au contrat d'insertion, aux contrats aidés ou aux contrats courts. C'est cette même logique de protection qui avait conduit le Gouvernement à rendre possible la validation de droits à la retraite de base au titre de l'activité partielle ou encore l'intéressement dans les entreprises de moins de onze salariés, de même que le maintien des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés en chômage partiel pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. La commission des affaires sociales du Sénat a introduit dans la loi la possibilité de déroger aux règles de cumul emploi-retraite que pratiquent les caisses de retraite en faveur des personnels soignants pendant la période épidémique. Le Gouvernement est favorable à cette mesure. Certaines dispositions dont l'urgence n'est pas totalement décorrélée de la crise du Covid-19 ont été placées au sein de l'article 2, ou transformées en articles additionnels, Elles sont relatives à l'indemnisation des victimes d'essais nucléaires, au statut des volontaires internationaux en ambassade ou encore à la gestion des fonds européens par les régions. Les incertitudes pesant sur le calendrier parlementaire nous ont conduits à privilégier ce vecteur pour vous les présenter. L'ordre du jour du mois de juin est particulièrement contraint. Il est soumis à l'évolution de la situation sanitaire. Des projets de loi électoraux vous seront vraisemblablement soumis, de même qu'un troisième PLFR qui comprendra d'importantes mesures de relance. Enfin, à l'automne, vous le savez comme moi, il n'y a guère de temps à consacrer à autre chose qu'au budget. Nous saisissons donc l'occasion de ce vecteur

L'article 3 visait à habiliter le Gouvernement à prescrire la centralisation du dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique et d'organismes privés chargés d'une mission de service public. Malgré la précision introduite par les groupes LaREM, MoDem et Les républicains à l'Assemblée nationale, qui a exclu de ce dispositif les organismes gérant un des régimes de retraite, la commission des finances du Sénat a supprimé cet article. Je comprends qu'il s'agit là avant tout d'une opposition à la méthode retenue par le Gouvernement plus qu'au fond de la mesure. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement propose que cet article soit rétabli. L'article 4 du projet de loi concerne le Brexit. Des explications plus approfondies vous seront données par ma collègue Amélie de Montchalin. Enfin, l'article 5 vise à prévoir un mécanisme de contrôle parlementaire des mesures réglementaires prises sur le fondement des habilitations prévues dans ce projet de loi. Après ces explications sur le fond des mesures présentées dans ce projet de loi, permettez-moi de dire quelques mots sur la méthode. Vous l'aurez compris, ce projet de loi concerne un très grand nombre de périmètres ministériels, ce qui n'était pas arrivé depuis les lois Warsmann de simplification du droit. C'est donc une chose assez rare et qui me permet, même si plusieurs de mes collègues nous rejoindront au cours des débats, de répondre au nom du Gouvernement à vos questions et à vos amendements. Nous Certains se sont émus et regretteront encore que ce projet de loi soit un texte « fourre-tout », selon l'expression qui a été utilisée en commission des lois. Mais je ne suis pas sûr que le dépôt de seize textes particuliers, soit autant de projets de loi que de périmètres ministériels, eût été préférable en termes de lisibilité De plus, et je m'exprime en tant que ministre chargé des relations avec le Parlement, organiser le calendrier d'examen de seize textes par l'Assemblée nationale et le Sénat eût été pour moi une véritable gageure S'agissant du recours aux habilitations, je n'ignore pas la sensibilité particulière qui s'attache au recours à l'article 38 de la Constitution. Je la comprends d'autant mieux que j'étais parlementaire- il pourrait m'advenir de le redevenir mais ce recours aux ordonnances est pleinement justifié par l'incertitude entourant l'évolution de la situation économique, sociale, sanitaire et administrative de notre pays à court terme. C'est sur ce fondement que le Conseil d'État, dans son avis rendu public, a validé le procédé. Le Gouvernement aurait pu se contenter, d'ailleurs, de mettre « en dur » les habilitations portant sur des dispositions législatives brèves et dont la rédaction est simple ou déjà avancée, comme l'y invitait le Conseil d'État. Il a pourtant veillé à aller plus loin, comme il s'y était engagé. Sur les 40 habilitations à légiférer par ordonnances, 16 ont été mises « en clair », si vous me permettez cette expression, à l'Assemblée nationale. Au stade de l'examen en commission, le Sénat a poursuivi ce travail précieux, puisque le projet de loi ne comporte plus que 10 habilitations, certes au prix de quelques suppressions, suppressions, s'agissant par exemple de l'article 3. Nous allons continuer ce travail en séance avec la transformation de l'habilitation sur la réserve civique, les instances consultatives des agences régionales de santé (ARS), le droit au chômage partiel des intermittents du spectacle, ou encore le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en position d'activité partielle. Le Gouvernement, conscient de la nécessité de préserver les droits du Parlement pendant la période de l'habilitation à légiférer par ordonnances, ne s'est pas opposé à la mise en place d'un dispositif de contrôle à l'article 5 du projet de loi. Certes, il demande que le délai prévu pour prendre les ordonnances prévues aux articles 1 et 2 soit à nouveau de six mois, et non pas de trois mois, comme vous le proposez. Ce délai est justifié, là encore, par l'incertitude entourant l'évolution économique dans les prochains mois et par le calendrier de négociation du futur budget européen. Je ne doute pas que nous aurons l'occasion de revenir plus précisément sur un certain nombre de ces points. Enfin, je n'ignore pas que ce projet de loi suscite des divergences entre le Gouvernement et votre assemblée. C'est d'ailleurs la vertu du débat parlementaire, auquel je suis, comme vous, très attaché. Je me réjouis de la qualité des travaux menés par vos commissions. Je voudrais saluer en particulier les trois rapporteurs, Mme Jourda, MM. Savary et de Montgolfier, qui ont chacun permis d'enrichir le texte et de confirmer sans les modifier plus de 13 dispositions votées par l'Assemblée nationale.

le projet de loi qui vous est soumis comporte des dispositions visant, comme vient de le dire Marc Fesneau, à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures nécessaires pour tirer les conséquences de la fin de la période de transition dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Avant d'en venir au détail des dispositions, je souhaiterais rappeler d'où nous venons et où nous souhaitons aller, car j'ai bien conscience de la difficulté que nous éprouvons tous à suivre le feuilleton du Brexit, qui dure maintenant depuis plus de trois ans. L'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, entré en vigueur le 1 février dernier, marque l'aboutissement de plus de deux ans de négociations difficiles conduites par le négociateur en chef au nom de l'Union, Michel Barnier. Cet accord préserve en particulier les droits acquis des citoyens britanniques et européens, notamment leurs conditions de séjour et de travail. C'était la première de nos priorités. Les citoyens français qui résidaient au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition pourront continuer à y vivre, travailler et étudier dans les mêmes conditions que celles qui prévalent actuellement. Réciproquement, les citoyens britanniques qui résidaient déjà sur le territoire français bénéficieront des mêmes droits qu'aujourd'hui. Notre mobilisation est totale pour la construction du futur partenariat avec le Royaume-Uni. Nous avons engagé le 2 mars dernier, le 2 mars dernier, toujours sous l'égide de Michel Barnier, une nouvelle négociation qui doit aboutir d'ici à la fin de la période de transition prévue par l'accord de retrait. Celle-ci doit s'achever le 31 décembre, mais elle peut être prolongée, à la demande du Royaume-Uni et avec l'accord de l'Union, d'un an ou de deux ans. Durant cette période de transition, l'accord de retrait prévoit que le droit de l'Union continue de s'appliquer au Royaume-Uni dans sa quasi-totalité. C'est un élément important de protection pour nos entreprises et nos concitoyens, qui permet de se préparer à une situation nécessairement différente de celle d'aujourd'hui. À la fin de cette période, seuls continueront en effet à s'appliquer l'accord de retrait et, si la négociation aboutit, l'accord sur la relation future. Notre objectif dans cette négociation est clair nous souhaitons conclure avec le Royaume-Uni un accord ambitieux et équilibré qui couvre un vaste champ- entre autres, le commerce, la pêche, les transports ou la sécurité -, tout en préservant les principes et les intérêts de l'Union. Construire une telle relation

les incertitudes n'ont jamais été aussi grandes, et d'abord sur le calendrier. Les Britanniques nous placent face à une contrainte de temps inédite pour négocier et ratifier l'ensemble du futur partenariat. Il nous reste désormais

de celui des Britanniques. Le défi est majeur, tant les sujets sont complexes et nombreux. À cela s'ajoute l'épidémie du coronavirus, qui nous a fait perdre un temps de négociation précieux,

la gouvernance de l'accord et les conditions de concurrence équitable. L'objectif demeure, Michel Barnier l'a confirmé, de tout faire pour défendre le mandat que les États membres lui ont confié le 25 février. Il est, selon nous, absolument inacceptable et hors de question

de nos agriculteurs, de nos entreprises, de nos concitoyens, sous prétexte de trouver un accord dans les délais et aux conditions imposés par les Britanniques. C'est pourquoi il est plus que jamais de notre devoir de nous préparer, de nous préparer, comme nous l'avions fait pendant la phase de négociation de l'accord de retrait, à tous les scénarios et en particulier à une absence d'accord à la fin de la période de transition. Tel est l'objet de la demande d'habilitation présentée par le Gouvernement à l'article 4 du présent projet de loi. Avant d'en venir au contenu des dispositions, je souhaite vous présenter l'approche que le Gouvernement a retenue pour cette demande d'habilitation. En premier lieu, le dispositif proposé se fonde sur le modèle, que vous connaissez, de ce que nous avions prévu dans le cadre de la loi d'habilitation de janvier 2019 pour préparer

retrait. Les dispositions qui vous sont proposées à l'article 4 permettent de traiter trois types de situations : d'abord, celles qui ne sont pas couvertes par l'accord de retrait ; ensuite, celles qui apparaîtraient en cas d'absence d'accord sur la relation future à l'issue de la période de transition, et qui sont du domaine bilatéral ; enfin, les situations particulières qui n'ont pas été identifiées jusqu'à présent, mais pourraient se présenter, et que nous envisageons par précaution dans le but de protéger nos concitoyens et les personnes qui se trouvent aujourd'hui sur notre sol. En tout état de cause, je tiens à le rappeler, la démarche de la France est pleinement respectueuse des compétences et des actions de l'Union européenne, dans le cadre de la négociation conduite au niveau européen. Les échanges que nous avons avec Michel Barnier sur ces dispositions sont, bien entendu, positifs, et nous n'entravons en sa capacité à négocier en notre nom. Certains sur ces travées- j'ai pu suivre vos échanges en commission -s'interrogent sur la nécessité de légiférer par ordonnances sur certaines de ces dispositions.

les personnes et les entreprises qui pourraient pâtir de l'effet couperet de la fin de la période de transition. Personne, je crois, ne peut contester ce besoin de protection. Le Parlement aura, bien sûr, l'occasion

Compte tenu de l'état d'avancement de la négociation, et en dépit du fait que les Britanniques s'y refusent pour le moment, personne ne peut exclure que cette période sera allongée. Il s'agit de trouver un juste équilibre entre les deux objectifs du Gouvernement limiter au maximum la période d'habilitation dans un esprit de consensus avec le Parlement et, d'autre part, maintenir une cohérence entre la négociation et la durée de la période de transition. Dans cet

Troisième point, nous vous demandons de nous permettre d'anticiper des problématiques ciblées dans une perspective de stabilité financière et de protection des assurés et des épargnants, et pour la bonne exécution des contrats

nous ne pouvons pas exclure aujourd'hui l'émergence de sujets résiduels, qui pourraient nécessiter une intervention au niveau national, mais qui, par définition, ne sont pas encore connus. Cette habilitation permettra, par exemple, à certaines professions soumises à des conditions d'exercice liées à l'appartenance à l'Union-

les sénateurs, nous sommes engagés dans une négociation sans précédent. Grâce à nos efforts collectifs et à votre soutien, nous avons franchi une première étape, celle de la sortie ordonnée du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le Gouvernement n'a pas eu besoin de faire usage de l'habilitation que vous lui aviez confiée en janvier 2019. 2019. Avec vous, je forme le voeu que nous puissions de nouveau trouver un accord ambitieux avec le Royaume-Uni d'ici à la fin de la période de transition, et que nous n'ayons pas à faire usage de l'habilitation que je vous demande de nous accorder aujourd'hui. Je le dis très solennellement, il faut nous préparer à toutes les éventualités

dans la mesure où le Parlement a toujours été présent et à la hauteur, me semble-t-il, des enjeux de cette crise. Il s'agit en effet du sixième projet de loi dont nous sommes saisis depuis le début de la crise sanitaire, deux projets de loi d'urgence, un projet de loi organique et deux projets de loi de finances rectificative. Parfois saisi de ces textes dans des conditions d'extrême rapidité,

est passé sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel précisément en raison des garanties qui avaient été introduites par le Sénat sur l'initiative de son rapporteur, qui n'est autre que le président de la commission des lois, Philippe Bas.

Deuxièmement, nous avons eu à coeur de vérifier que les habilitations demandées étaient précises. Lorsque le Parlement se dessaisit de ses pouvoirs, il doit en effet savoir

Un principe : légiférer dans l'urgence, certes, mais pas au-delà de ce que commande la situation de crise, et dans la mesure du possible en toute connaissance de cause. Il faut bien reconnaître qu'un qu'un certain nombre d'études d'impact manquaient au dispositif. Nous avons donc exclu les habilitations trop larges, les dispositifspermanents et les chiffrages

projet de loi habilite le Gouvernement à prévoir des règles différentes d'un secteur à l'autre, afin de cibler au mieux le soutien public sur les entreprises les plus en difficulté. même celles qui ne connaissent pas de gros problèmes devront continuer à être encadrées. En revanche, les paramètres d'indemnisation des salariés en activité partielle et de remboursement

juin. Les différents amendements que nous examinerons et qui tendent à reporter dans le temps la possibilité pour le Gouvernement d'adapter ces règles relatives à l'activité partielle n'atteindront peut-être pas l'objectif recherché par leurs auteurs. Nous aurons l'occasion d'en discuter. Il faut permettre une adaptation à plusieurs vitesses du dispositif, en fonction de la situation et descaractéristiques des entreprises, de manière à inciter à un retour à l'activité très important tout en limitant les impacts sociaux

paramètres qu'il est envisagé de modifier, et surtout sur l'impact attendu de ces mesures. Nous attendons des précisions de la part du Gouvernement. l'initiative de la commission des affaires sociales, plusieurs habilitations en matière de droit du travail ont été inscrites en clair dans le projet de loi, concernant l'indemnisation du chômage, la représentation des travailleurs indépendants, le prêt de main-d'oeuvre, ainsi que, conjointement avec la commission des lois, le mandat des conseillers prud'hommes et la représentation des salariés des TPE. Ces mesures, le plus souvent ponctuelles, ne justifiaient pas une habilitation à légiférer par ordonnance. La commission s'est par ailleurs attachée à clarifier la rédaction des articles visant à assouplir les règles relatives aux contrats courts, d'une part, et aux contrats d'insertion et contrats aidés, d'autre part, en veillant notamment à bien limiter dans le temps la possibilité de déroger par accord d'entreprise aux règles de renouvellement des CDD.

aides, au vu du contexte exceptionnel que nous connaissons, la commission a validé une situation de fait, l'aide de 1 milliard d'euros ayant déjà été versée et financée sur les réserves du régime complémentaire des indépendants, et destinée aux artisans et commerçants Nous avons d'ailleurs laissé cette souplesse, également, pour les caisses complémentaires, comme celles des professions libérales, notamment des avocats. Le second point concerne la validation des périodes d'activité partielle au titre de la durée d'assurance permettant l'ouverture des droits à la retraite. La commission a choisi de limiter strictement le champ du dispositif

loi pour prescrire le dépôt, sur les comptes du Trésor, des disponibilités non seulement des personnes morales soumises aux obligations de la comptabilité publique, mais également des organismes publics ou privés chargés d'une mission de service public.

que la direction générale des finances publiques ne pourraient leur fournir. En outre, la centralisation des dépôts me semble présenter un certain nombre d'avantages, en matière de gestion des deniers publics, notamment celui de réduire le coût des émissions de titres de financement

elle ne valide la méthode employée par le Gouvernement pour introduire ce dispositif dans le projet de loi. Tout d'abord- cela a été dit par Muriel Jourda -, le champ de l'habilitation est beaucoup trop large, puisqu'il fait référence aux « organismes publics ou privés chargés d'une mission de service public

il me semble prématuré d'inscrire ces dispositions dans le présent projet de loi, puisque, manifestement, le Gouvernement n'a pas encore commencé les concertations indispensables avec les différents organismes.

Oui, la démocratie doit reprendre tous ses droits et, en l'espèce, la démocratie parlementaire aussi. Or ce n'est pas l'image donnée par ce texte, qui se prive ainsi des conditions de la confiance. Les crises ont un pouvoir révélateur, du meilleur comme du pire. Cette crise épidémique donne une image crue de la pratique de votre pouvoir,

Pourtant, même et surtout en temps de crise, le Parlement est bien, au sens étymologique du terme, l'endroit où l'on parle. Dans cette enceinte, on débat pour faire la loi, l'expression de la volonté générale à laquelle tous les citoyens ont le droit de concourir, personnellement ou par leurs représentants. En définitive, sur quoi, dans ce texte, les parlementaires seraient-ils autorisés à parler, donc à légiférer ? était, initialement, truffé de 40 demandes d'habilitation à légiférer par ordonnance ; ce recours massif ne relève pas uniquement de l'urgence, il traduit à l'envi le refus du débat contradictoire par le Gouvernement. 40 habilitations se seraient ajoutées aux précédentes, dont on verra si la ratification est inscrite à l'ordre du jour. Chaque alinéa de ce texte était donc un blanc-seing ; chaque article était un cavalier législatif, dont le caractère urgent était plus que relatif. Si certaines habilitations sont directement liées à la crise, d'autres viennent tout simplement pallier le retard pris par le Gouvernement- c'est le cas pour ce qui concerne le code de la justice pénale des mineurs -ou servent à recycler des dispositions insérées dans des textes en cours de navette. C'est, en méprisant, la plupart du temps, les travaux du Sénat. Ainsi, dans cette enceinte où l'on parle, nous serions surtout autorisés par ce gouvernement à nous taire Faut-il le rappeler, l'habilitation n'est pas une délégation du pouvoir législatif : le Parlement conserve, avec le référendum, le monopole de faire la loi. Il s'agit juste d'une extension momentanée du pouvoir réglementaire ; il faut constamment le garder à l'esprit. les délais d'habilitation à légiférer retenus par le Gouvernement dans ce texte étaient anormalement longs pour des mesures dites « d'urgence ». Par ailleurs, Guy Carcassonne je ne peux que citer sa pensée -, les ordonnances ont souvent « rendu un [ ...] grand service : [elles ont] prouvé que [ ...], pour faire de bonnes lois, on n'a pas encore inventé mieux que le Parlement. Les ordonnances [ ...] sont [ ...] comme des projets qui deviendraient directement des lois. Ce sont généralement des textes défectueux, dont les malfaçons ne se révèlent qu', là où se serait sans doute trouvé un parlementaire pour soulever,

Malgré ce « tamis parlementaire », ce texte demeure comme la créature de Frankenstein : les juxtapositions ne lui donnent pas vraiment de corps. Par ailleurs, son absence de ligne directrice et de cohérence complexifie son examen. le Gouvernement fait la preuve de la mauvaise qualité initiale du texte : il dépose des amendements de séance kilométriques et en quantité industrielle- non moins de 30 amendements sur un texte qui contenait, je le rappelle, 4 articles -, ajoutant encore-

Or mal légiférer parce que le texte initial est médiocre et parce que les conditions ne sont pas réunies pour son bon examen, c'est nuire à la qualité de la loi, qui touche le quotidien des Français ; donc c'est nuire au quotidien des Français. En définitive, la pratique actuelle de l'exécutif, même si elle a pu, initialement, se justifier, n'est que l'exacerbation de sa pratique antérieure, fondée sur une pensée teintée de libéralisme : la concentration du

texte fourre-tout, qui noie le Parlement, tout en glissant çà et là une nouvelle dose de dérégulation du droit social, texte troué par des ordonnances et même refus de consultation quand la démocratie sociale est jugée superflue, ce dont s'offusque même le Conseil d'État.

n'autorise pas le dessaisissement du Parlement, même si la tentation des pleins pouvoirs est forte sous la V République. Puisque, comparativement à d'autres, notre Parlement est l'un des plus faibles parmi les démocraties occidentales, il faut que les pratiques gouvernementales ne le dessaisissent pas encore un peu plus. Le

plus. Petit à petit, un phénomène d'accoutumance à la marginalisation du Parlement s'installe : ce qui était l'exception devient la règle et l'anormalité devient une nouvelle normalité. Comme s'il était contaminé, lui aussi, par un étrange virus, le Parlement s'atrophie. C'était d'ailleurs la perspective de votre révision constitutionnelle. Or, quand le Parlement est malmené, c'est la démocratie qui s'abîme. Il y a, dans l'histoire, des contrastes. Certains ont récemment tissé une métaphore martiale autour de la période exceptionnelle que nous vivions. Soit, mais, en temps de guerre, le Parlement n'a pas toujours été marginalisé, voire muselé.

parlementaire, maintenir les prérogatives du Parlement. Chacune de ses décisions était soumise à débat. Comme le disait André Pierre, il voulait apporter à l'Angleterre et au monde la preuve que l'on pouvait faire la guerre et vaincre sans porter atteinte aux libertés du peuple et que le courant de confiance mutuelle existant entre le Gouvernement et les élus de la Nation était l'un des plus sûrs garants de la victoire.

Parce que nous sommes plus qu'attachés aux droits du Parlement, en ce qu'ils garantissent la délibération, le débat, la contradiction, nous lançons une alerte et nous demandons le rejet de ce texte, au travers de l'adoption de cette motion tendant à opposer la question préalable. La crise sociale sans précédent que nous traversons, que nous devrons surmonter, trouvera ses solutions non dans la verticalité, dans la mise en sourdine du Parlement, mais dans la vitalité démocratique, dans la dialectique des chambres, dans la consultation des corps intermédiaires. C'est une question de confiance. Jamais Créon ne pourra gouverner sans Antigone. Vous avez raison, monsieur le ministre, oui, il est temps que la démocratie reprenne tous ses droits

que le Gouvernement peut demander au Parlement de l'habiliter à prendre, par ordonnances, des mesures législatives. Le mot « programme » n'est pas dénué de portée dans la Constitution, car on le retrouve dans l'une des dispositions les plus importantes

longuement hésité avant de prendre la parole pour m'opposer à votre motion, mes chers collègues. En effet, tout aurait dû m'orienter vers cette solution. Néanmoins, dans un instant de raison, je me suis dit que, si nous adoptions votre motion, alors le Gouvernement, dans un dialogue singulier avec l'Assemblée nationale- dialogue qui ressemble parfois à une sorte de monologue à plusieurs voix, si l'on peut s'exprimer ainsi

que celui que nous espérons imposer, au travers d'un rapport de force entre les deux assemblées. Cela s'appelle le bicamérisme. vous êtes entré dans cet exercice parlementaire avec 37 habilitations ; l'Assemblée nationale les a elle-même ramenées à 24 ; notre rapporteur s'apprête à vous proposer de les faire descendre à 10.

adoptons-les, tout en gardant un droit de regard et en faisant en sorte que leur durée soit limitée et que le Gouvernement ait à revenir devant le Parlement chaque fois qu'il aura besoin de nouveaux pouvoirs lui soient conférés. C'est la raison pour laquelle la commission des lois et son rapporteur, qui m'a autorisé exceptionnellement à prendre la parole, à condition que je n'en abuse pas- peut-être est-ce malheureusement déjà le cas

disons-le d'emblée, ce projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ne nous convient pas. tout d'abord, la méthode. Voilà des mois que le Gouvernement veut un Parlement aux ordres : systématisation de la procédure accélérée, recours massif aux ordonnances, conditions déplorables Avec l'état d'urgence sanitaire, ces mauvaises pratiques se sont encore amplifiées. Certes, la crise sanitaire, économique et sociale nécessite d'agir vite, mais pas au prix du mépris du Parlement. Monsieur le ministre, vous qui êtes chargé des relations avec le Parlement, sachez que nous n'acceptons pas d'être dessaisis de notre capacité de faire la loi ; nous n'acceptons pas de nous satisfaire d'une habilitation puis d'une loi de ratification que, la plupart du temps, nous attendons longtemps ; nous n'acceptons pas qu'il ne nous reste qu'à « encadrer » des ordonnances et à vous laisser gouverner seuls. seuls. Nous ne nous habituons pas à ce que vous confiniez le Parlement ; nous sommes là pour faire la loi, pour la nourrir, par le dialogue et l'échange, et pour agir en responsabilité. Avec ce texte, vous nous livrez la quintessence de votre conception du travail parlementaire : à l'origine, le projet de loi ne contenait pas moins d'une quarantaine de demandes d'habilitation. Le Conseil d'État s'en est ému et l'Assemblée nationale, suivant l'avis de cette Sans colonne vertébrale, sans lien entre les articles, ce texte est un fourre-tout, un salmigondis, un enchaînement de cavaliers législatifs dont l'essentiel n'a pas de lien avec la crise sanitaire. Quel rapport entre la justice des mineurs, les chèques-restaurant, les victimes des essais nucléaires, les volontaires internationaux, la situation des doctorants, la réglementation des ventes à perte ou encore le Brexit ? Un véritable inventaire à la Prévert La commission des lois du Sénat a fait, comme à l'accoutumée, son travail avec sérieux. Je salue les options proposées par sa rapporteure pour ramener le nombre des habilitations à 10, pour réduire la durée de celles-ci, pour transposer certaines dispositions dans le dur de la loi et pour supprimer un certain nombre de dispositions. je souligne l'initiative unanime de la commission des finances de proposer la suppression de l'article 3, par lequel le Gouvernement s'apprêtait à faire main basse sur la trésorerie de toute une série d'institutions, dont on ne connaît d'ailleurs même pas la liste. Si, sur la forme, les avancées sont significatives, nous regrettons que la commission ne nous ait pas suivis sur le fond, car l'esprit de ce texte reste préoccupant. Au détour de mesures anecdotiques se tapissent un certain nombre de mauvais coups, avec, je le regrette, l'assentiment de la majorité sénatoriale.

Autre exemple, pour répondre au besoin de main-d'oeuvre agricole, le Gouvernement porte la durée de séjour des travailleurs saisonniers étrangers de six à neuf mois, mais sans droits nouveaux, et il autorise les étudiants étrangers à travailler jusqu'à 80 % du temps sans prévention pour la qualité de leurs études. Voilà une main-d'oeuvre bon marché vous appelez cela « pragmatisme » ; nous répondons : « utilitarisme » ! Dernier exemple- nous aurons l'occasion d'en citer d'autres -, l'utilisation des volontaires internationaux pour remédier aux lacunes en ressources humaines du ministère des affaires étrangères. D'autres sujets nous préoccupent, notamment en matière de justice, comme l'extension de l'expérimentation des cours criminelles sans évaluation ni recul, alors que, dans le même texte, on souhaite mobiliser plus de jurys populaires. De même, nous nous inquiétons de l'absence de débat parlementaire sur la réforme de la justice des mineurs et du report de sa mise en oeuvre. Enfin, nous proposons de supprimer l'article 4 relatif aux conséquences du Brexit, considérant que ce sujet nécessite à lui seul un débat approfondi et plus large que les seuls sujets abordés dans ce texte, dès que le Royaume-Uni aura fait connaître, le 1 juillet prochain, son intention de prolonger ou non la période de transition. Monsieur le ministre, ce texte, que vous aviez intitulé, à l'origine, « projet de loi portant diverses dispositions urgentes » n'a rien d'un texte d'urgence pour répondre aux conséquences de la crise du Covid-19.

soutien aux collectivités locales, sécurisation des parcours d'insertion, maintien du versement des pensions alimentaires par les CAF, etc. Nous regrettons que la commission ait, une fois de plus, fait un usage extensif de l'article 45 de la Constitution, nous privant d'un débat sur bon nombre de ces sujets. Monsieur le ministre, pour nous, l'urgence est sociale. Ce projet de loi est malheureusement vide de mesures pour y répondre. La parole président, monsieur le ministre, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, vous pardonnerez autant que vous comprendrez, je l'espère, que je revienne sur la forme de ce projet de loi, celle-ci étant indissociable de son fond. Ce texte se présente à l'évidence comme une compilation de dispositions disparates, qui visent largement à habiliter le Gouvernement à prendre des ordonnances dans les domaines les plus divers. Les conséquences du Brexit côtoient les contrats de travail, et les pouvoirs des fédérations sportives les titres-restaurant, pour ne citer que ces quelques exemples. Cela a déjà été dit, mais il faut bien y revenir, la cohérence et la clarté qui manquent à ce projet de loi ont des conséquences directes sur la qualité de la délibération parlementaire. Si l'on y ajoute les délais d'examen du texte- un problème que le seul contexte sanitaire ne saurait justifier -, on ne peut s'empêcher de penser que ce projet de loi condense en lui-même tous les défauts que l'on adresse couramment aux évolutions, néfastes, de la procédure législative : recours quasi systématique à la procédure accélérée, délai pour le dépôt des amendements incompatible avec une réflexion poussée, habitude de légiférer par ordonnances, pratique malheureuse des lois fourre-tout, qui évoque le triste souvenir des lois Warsmann. Les conditions extrêmes d'examen de la loi du 11 mai dernier n'ont apparemment pas permis d'inverser la donne. Bien sûr, les circonstances actuelles exigent certains accommodements. Nous en convenons tous. Aussi le Sénat a-t-il réorganisé ses travaux comme l'imposait la crise sanitaire, mais les modalités d'examen de ce projet de loi traduisent une forme de déconsidération et ne doivent en aucun cas constituer un précédent. Pour toutes ces raisons, il est malaisé de se forger une opinion aboutie sur ce texte. Puisqu'il m'est impossible d'en traiter dans ses détails comme dans sa globalité, je ne relèverai que quelques points saillants. Concernant les conséquences de la crise sanitaire, nous nous réjouissons des dispositions qui protègent ceux qui en ont le plus souffert, par l'incertitude qui plane désormais sur leur situation ou la précarité qui les touche. La prolongation des titres de séjour, le maintien des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés en activité partielle et l'adaptation des règles relatives aux contrats d'insertion s'inscrivent tous dans cette lignée. Nous nous en félicitons. Il en va également ainsi de la mobilisation des réserves des caisses complémentaires des indépendants, de la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à la retraite et de la dérogation aux règles de cumul emploi-retraite pour les soignants. Les conséquences que cette crise emporte sont multiples et probablement, pour certaines, encore inconnues. Il est heureux que l'action de l'État réduise ses effets néfastes, en s'adaptant dans chaque domaine. Je pense particulièrement au fonds de soutien aux restaurateurs et à la singularité de son mode de financement. Il importe cependant de veiller à ce que certains remèdes ne s'inscrivent pas dans le droit commun. Il est raisonnable que les circonstances actuelles, qui conjuguent incertitude et nécessité d'une reprise économique, exigent une adaptation par accord d'entreprise des règles relatives aux contrats courts, mais il serait regrettable que celle-ci devienne la norme. C'est à raison que la commission des affaires sociales du Sénat a prévenu un tel glissement, en fixant un terme à son application. Concernant l'habilitation relative au Brexit, on ne peut, en premier lieu, que se satisfaire de la réduction de sa durée d'application. Il faut observer, dans un second temps, que, si la plupart des domaines en cause relèvent de questions techniques qui justifient, compte tenu de l'urgence, le recours aux ordonnances, ce n'est pas le cas de tous. Le maintien des licences et des autorisations de transfert vers le Royaume-Uni de produits et matériels de défense comme les problèmes que soulèvent certains contrats d'assurance et plans d'épargne en actions demandent une solution juridique pour laquelle les ordonnances sont adaptées. En revanche, la désignation de l'autorité nationale chargée de la sécurité du tunnel sous la Manche et la définition du régime des ressortissants britanniques sur le territoire national ne justifient en rien une telle habilitation. là se priver inutilement des vertus de la délibération parlementaire. Enfin, le groupe RDSE soutient les amendements que Mme la rapporteure de notre commission des lois a apportés au texte la réduction du délai d'habilitation, la suppression d'un potentiel effet rétroactif et l'amélioration du dispositif d'information des parlementaires garantissent à raison le bon exercice par les chambres de leur mission constitutionnelle de contrôle. Il en va également de la sécurité juridique de notre droit, principe qui a été éprouvé au cours des derniers mois et qu'il nous importe de réhabiliter au mieux et au plus vite. La qualité de la loi dépend de celle du dialogue entre le Gouvernement et le Parlement. Plus qu'une question de légistique ou une observation pratique, c'est un impératif démocratique. C'est pour cette raison que le groupe RDSE sera très attentif aux débats, qui lui permettront d'éclairer son jugement et de décider de son vote. Nous devons dès maintenant poser les premiers jalons de la méthode que nous appliquerons pour conduire l'action de l'État dans la gestion d'une crise qui survivra à son volet sanitaire. La transparence, le dialogue institutionnel et la délibération parlementaire sont des éléments essentiels, voire tout bonnement nécessaires à la réussite de toute politique. La parole Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, notre pays traverse depuis plus de deux mois une crise sanitaire sans précédent, qui a des conséquences considérables et diverses en matière économique, sociale, administrative et sanitaire. C'est la raison pour laquelle, ces dernières semaines, nous avons été appelés, pour y faire face, à effectuer les aménagements nécessaires à notre cadre juridique, au travers de l'examen et du vote de plusieurs projets de loi. Nous sommes aujourd'hui de nouveau réunis pour nous prononcer sur une série de mesures qui viendront compléter ces dispositifs. Sur la forme, il est vrai que les délais d'examen ont été courts. Comme l'ensemble des Français, nous privilégions autant que faire se peut le télétravail, ce qui complexifie notre activité, celle de l'administration du Sénat et de nos collaborateurs, mais l'urgence de la situation et son caractère inédit commandent que l'on légifère plus rapidement et que l'on adapte nos conditions de travail. Nous sommes en capacité de le faire. Par ailleurs, ce texte contenait initialement un certain nombre- pour ne pas dire un nombre certain - d'habilitations à légiférer par ordonnances. Comme tout parlementaire, je n'en suis pas friand, même si je reconnais que le recours aux ordonnances peut s'avérer utile lorsqu'il est mû par l'urgence et la technicité des mesures.

Le Conseil d'État s'était prononcé en faveur d'une telle démarche pour les dispositions brèves dont la rédaction était simple ou déjà très avancée ; le Gouvernement comme le Parlement ont épousé cette voie. Ce travail devrait se poursuivre aujourd'hui en séance, dans une démarche commune de clarification que nous pouvons saluer. Pour finir sur les débats de forme, il me semble important de rappeler que le contrôle du Parlement sur la préparation et la mise en oeuvre des quelques ordonnances restantes, introduit à l'Assemblée nationale et dont la rédaction a été précisée par le Sénat, permettra d'achever de rassurer ceux qui craignent un hold-up démocratique. Le rôle du Parlement a bien été préservé. J'en au fond du texte. Certains ont qualifié ce projet de loi de « fourre-tout ». Je retiendrai, pour ma part, un texte très dense, certes, mais qui se justifie par la multitude des secteurs touchés. Il vient répondre à plusieurs attentes de la population, exposée à des difficultés économiques et à des incertitudes sur l'avenir, et accompagne les conditions d'une relance de l'activité. Je pense aux droits à la retraite au titre des périodes d'activité partielle. Notre groupe a d'ailleurs déposé un amendement sur ce sujet, afin de revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale, qui nous semble plus protectrice. Je pense également à l'augmentation de la durée de travail annuel maximale autorisée pour les étudiants étrangers, à la sécurisation des parcours d'insertion ou encore à la neutralisation de l'effet de la crise sanitaire sur la transformation des CDD en CDI dans la fonction publique.

En tant que commissaire aux lois, je ne peux pas ne pas m'arrêter un instant sur les dispositions relatives au fonctionnement de la justice. Des réserves ont été émises en commission sur l'extension à trente départements de l'expérimentation de la cour criminelle. Elles s'expliquent par la sensibilité de ces sujets, confrontée aux incertitudes liées à la période particulière de crise que nous continuons à traverser.

Je veux également saluer le report opportun de l'entrée en vigueur de plusieurs réformes civiles et pénales, qui n'a pas été remis en cause par la commission. Il devrait notamment permettre à l'autorité judiciaire d'être prête pour l'application de réformes indispensables et à notre Haute Assemblée de pouvoir mener, dans des délais raisonnables, le débat parlementaire envisagé sur le nouveau code de la justice pénale des mineurs. Les auditions ont d'ailleurs commencé, monsieur le président de la commission des lois. Je veux enfin saluer les dispositions relatives aux territoires d'outre-mer, qui n'auraient pas trouvé rapidement de véhicules législatifs dans lesquels s'insérer, alors même qu'elles sont très attendues localement. Je pense à la prolongation d'un an de l'activité des agences des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe et de la Martinique et, par conséquent, au report du transfert des espaces concernés aux collectivités territoriales. Je pense également à la prolongation de deux ans de l'activité de la commission d'urgence foncière de Mayotte, chargée d'aider les particuliers dans leurs démarches de régularisation foncière, avant qu'elle ne soit transformée en groupement d'intérêt public. Pour compléter ces adaptations particulièrement bienvenues, nous présenterons tout tout à l'heure un amendement qui permet de maintenir l'échéance de la création du conseil de prud'hommes de Mayotte. Mes chers collègues, je crois sincèrement que le texte dont nous débattons aujourd'hui a fait et continuera de faire l'objet d'un travail de réflexion commune, dans une démarche de clarification partagée,

notamment s'agissant du Brexit. Les délais ont été jugés trop longs et contradictoires avec l'urgence du projet de loi. J'attire cependant votre attention sur le fait que nous n'avons absolument aucune visibilité quant à la reprise d'une activité « normale Ce temps supplémentaire permettrait de tenir compte de cet état de fait, pour une meilleure organisation du travail du Gouvernement, face, notamment, concernant les mesures relatives au Brexit, à l'incertitude profonde sur la durée de la période de transition. Nous en débattrons dans les prochaines heures. Nous aurons également à débattre de la centralisation des trésoreries publiques, qui permettrait de réduire l'endettement et l'appel aux marchés de l'État, dans un contexte de forte sollicitation du Trésor. Je veux croire, mes chers collègues, que notre Haute Assemblée saura dépasser ces divergences, afin d'avancer sur des sujets essentiels pour accompagner la reprise, dans l'intérêt de notre pays. La parole

Cette demande d'habilitation pose problème, car elle élargit l'obligation de dépôt au Trésor public pour plusieurs organismes, particulièrement les collectivités territoriales. Or, en transférant leurs trésoreries sur le compte du Trésor public, non seulement celles-ci perdront une autonomie de gestion, mais elles seront également privées des ressources financières procurées par les intérêts. Par ailleurs, cette centralisation s'appliquerait aussi aux organismes chargés d'une mission de service public, notamment ceux qui interviennent dans des secteurs essentiels tels que le transport, l'eau, l'énergie ou l'assainissement. Le moment est mal choisi pour les priver d'une gestion autonome, qui leur permet d'agir de manière plus souple et de déployer des capacités d'investissement plus que jamais nécessaires. Dans la crise que nous traversons actuellement, cette perte de recettes constituerait un frein supplémentaire à l'autonomie fiscale des collectivités. Elle viendrait s'ajouter- faut-il le rappeler -à la baisse continue des dotations de l'État et à la suppression récente de la taxe d'habitation. Enfin, les pertes budgétaires ont encore été alourdies par la gestion de l'épidémie du Covid-19, qui a entraîné des coûts supplémentaires imprévus. Un tel contexte ne peut que fragiliser les collectivités, au moment où elles ont un rôle majeur à jouer dans le soutien et la relance du tissu économique local. Pour toutes ces raisons, je soutiens sans réserve la suppression de l'article 3, adoptée dans le texte de la commission des lois. C'est une condition indispensable de l'adoption de ce projet de loi.

Vous demandez au Parlement une délégation de son pouvoir législatif dans des domaines aussi variés que le droit social, le droit de la consommation, les finances publiques, le droit pénal, le droit d'asile, le droit européen, le code de la défense, le code de l'environnement, sans lien avec la gestion de la pandémie, aux seules fins de faire l'économie d'un débat de fond et d'éviter d'avoir à justifier vos choix devant les députés et les sénateurs. Dans sa version initiale, ce projet de loi prévoyait 40 ordonnances, que le Gouvernement entendait prendre dans un temps extrêmement resserré, faisant fi du principe constitutionnel de clarté de l'élaboration de la loi. La seule ligne directrice de ce texte sans cohérence est de pallier le retard pris par le Gouvernement en amont de la crise sanitaire, reprenant des dispositions éparses de textes en cours de navette parlementaire. Comment pourrions-nous accepter, en cette période d'incertitude et d'inquiétude, en cette période de défiance profonde de la population à l'égard de l'exécutif, le blanc-seing que vous demandez, alors qu'une cinquantaine d'ordonnances plus anciennes doivent encore être ratifiées ? Comment pourrions-nous accepter l'instrumentalisation de l'urgence sanitaire pour nous départir de notre pouvoir législatif pour un temps anormalement long, les délais des habilitations prévues initialement variant entre six et quinze mois à compter de la publication de la loi ? Nous saluons, à cet égard, le travail de la commission des lois, qui a réduit le champ et la durée de nombreuses ordonnances et qui a rappelé que le Gouvernement devrait présenter les projets de loi de ratification de ces dernières dans un délai de deux mois. Comment accepter que, dans ce brouillard législatif, le Gouvernement puisse profiter de la confusion et de l'inquiétude générale pour prendre des mesures qui vont nuire aux Français ? Ne nous y trompons pas : si certaines mesures sont directement liées à l'épidémie de Covid-19- il y va ainsi des règles applicables au chômage partiel, de la fin anticipée des saisons sportives, de la prolongation du versement de l'allocation pour les demandeurs d'asile et des contrats aidés -, d'autres, en revanche, et non des moindres, sont des attaques en règle contre le droit du travail ou le pouvoir judiciaire, ou encore en faveur d'intérêts particuliers, voire purement électoraux. Pour illustrer mon propos, quelle urgence y a-t-il à favoriser l'ouverture de la saison de la chasse, alors que nos concitoyens sont encore limités dans leur liberté d'aller et venir et doivent se soumettre aux gestes barrières afin d'éviter une seconde vague ? Que dire de la possibilité laissée aux employeurs de multiplier les contrats à durée déterminée hors de toute contrainte et de déroger au nombre de vacations dans toute une série de missions publiques ? ? Nous le savons, l'assouplissement des règles relatives au CDD et à l'intérim s'est toujours accompagné d'une précarisation des conditions d'emploi pour les travailleurs concernés, sans effet significatif en termes de relance économique, d'autant que cette mesure a été aggravée par la commission des affaires sociales, qui ne souhaitait pas que les dérogations aux règles de renouvellement des soient neutralisées par la durée de trente-six mois prévue à l'article 1 A. Il s'agit des contrats conclus dans le cadre des parcours emploi compétences, en particulier des contrats uniques d'insertion. Quelle urgence y avait-il à inscrire dans ce texte une mesure du projet de loi ASAP permettant aux entreprises de moins de onze salariés de mettre en place un dispositif d'intéressement par décision unilatérale de l'employeur et de prévoir sa reconduction tacite, alors que, dans le même temps, nous savons que de nombreuses familles risquent de voir leurs revenus diminuer à partir de juin si les enfants ne retournent pas à l'école à l'école ? Que dire encore de l'allongement de la durée de séjour des travailleurs étrangers afin de disposer d'une main-d'oeuvre peu contraignante et corvéable à merci ? Si la mesure est de bon sens, rien n'est prévu sur leurs conditions de travail et de rémunération. Or il semble que les contraintes sanitaires renforceront le caractère inacceptable des conditions de travail de ces travailleurs, pourtant essentiels. Dans le même temps, rien ou presque n'est prévu pour les travailleurs saisonniers. La plupart de ces affaiblissements pourront se prolonger plusieurs mois après la fin de l'état d'urgence. Au lieu de proposer un grand plan de relance, avec des droits sociaux nouveaux et des filets de sécurité pour tous, ce texte ne fait qu'étendre la précarité et la casse des conquis sociaux. De même, comment justifier l'élargissement de l'expérimentation des cours criminelles- rejeté en commission -, à rebours des engagements pris par le Gouvernement au moment du débat sur la réforme de la justice ? Malgré le travail sénatorial et la réduction du nombre d'habilitations de 24 à 10, le recours aux ordonnances participe de la dégradation du Parlement. Cela n'est pas acceptable. Le Parlement n'est pas une institution qu'il faudrait occuper afin de se donner bonne figure. Dans cette période d'entre-deux, entre confinement et perspectives de déconfinement total, nous refusons d'être infantilisés et revendiquons le respect de notre légitimité démocratique. Renoncer encore et toujours à nos compétences, c'est oublier que le mandat qui nous a été confié par les Françaises et les Français doit être respecté. C'est oublier que, si, à l'instar de la vie économique, sociale et culturelle, la démocratie a été percutée de plein fouet par la crise que le pays traverse, elle doit rester debout, ne pas être malmenée, bafouée, bâillonnée, sous peine de faire violence aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, auxquelles nous sommes très majoritairement ici attachés. L'urgence ne justifie pas la précipitation. Elle ne justifie pas que le Parlement soit entravé dans sa capacité d'analyse et de décision éclairée. C'est pourquoi nous voterons contre ce projet de loi, qui n'a d'urgent que le titre.

ces dernières semaines ont mis un coup d'arrêt à notre économie. Notre PIB s'est contracté de 5,8 % au premier trimestre, un record depuis 1949. Nous savons que nous allons devoir faire face, dans les prochains mois, à une crise économique d'une ampleur considérable et préoccupante. Nous devons l'anticiper et nous y préparer. Ce texte que nous examinons comporte plusieurs mesures en ce sens. Il s'agit d'assurer la pérennité des entreprises fragilisées par la crise. Pour cela, l'État a largement activé le régime de chômage partiel, permettant de mettre en sommeil bon nombre d'entre elles. L'économie redémarre doucement, sans doute trop lentement encore et, pour l'accompagner, nous devons apporter aux entreprises la flexibilité dont elles ont besoin. Le confinement a engendré d'importantes pertes d'activités qui ne sont pas sans conséquences sur les contrats de travail. Dans les six prochains mois, les CDD, les contrats de mission ou encore les contrats uniques d'insertion pourront être conclus ou renouvelés pendant une durée de trente-six mois, contre vingt-quatre mois auparavant. Il faudra cependant les encadrer par des accords d'entreprise et, bien évidemment, comme c'est prévu dans le texte, les limiter dans le temps. Autre mesure à destination des TPE, un régime d'intéressement pourra être mis en place pour une durée maximale de trois ans. Le groupe Les Indépendants croit beaucoup à l'intéressement, qui lie l'intérêt des entreprises à celui des salariés. C'est, à nos yeux, un dispositif juste, qui permet de partager le fruit de l'activité avec ceux qui contribuent à la faire naître. Cette mesure contribuera aussi à relancer l'économie. Toutefois, avant de parler d'intéressement, il faut préalablement qu'il y ait création de richesses. À cet égard, notre groupe voulait proposer (EPCI), déjà très mobilisés en faveur des entreprises de leur territoire, puissent octroyer et gérer eux-mêmes les aides aux entreprises en difficulté, bien évidemment en complémentarité avec les régions.

Il est aussi prévu que les salariés concernés par une activité partielle disposeront des mêmes droits à la retraite que s'ils avaient été employés à plein temps. C'est là une mesure importante dans le contexte actuel. Le secteur privé n'est pas le seul à devoir s'adapter aux circonstances exceptionnelles de cette crise que nous traversons. La fonction publique a elle aussi besoin de souplesse. Ainsi, les militaires et les chercheurs pourront voir leurs droits et contrats prolongés. Par ailleurs, nous nous félicitons des dispositifs permettant le cumul des pensions civiles et militaires avec les revenus liés aux activités dans les hôpitaux publics et privés, au plus fort de la crise. C'est bien là le minimum que nous devions à toutes celles et à tous ceux qui se sont mis au service de la santé de nos concitoyens durant le pic de l'épidémie. La situation des travailleurs étrangers en France a aussi été impactée par la pandémie. Elle a besoin d'être clarifiée. Le plafond d'activité des travailleurs saisonniers étrangers présents en France au 16 mars sera relevé de six à neuf mois

au secteur agricole, déjà très fragilisé avant cette crise et encore plus aujourd'hui. Les étudiants étrangers seront également autorisés à travailler de manière dérogatoire- jusqu'à 80 % -, en attendant la reprise effective des cours. Tout comme l'économie, l'ensemble de l'activité sociale doit reprendre. C'est absolument indispensable. Je pense notamment à la justice. Le retard accumulé en la matière est considérable. Pour faire face à cet afflux, les tribunaux vont devoir employer des moyens exceptionnels. Nous souhaitons cependant que cela ne nuise pas au respect des règles et des procédures les plus élémentaires, en particulier au tirage au sort des jurés d'assises. Il est impératif que le public puisse assister Nous vous proposerons de voter des amendements en ce sens, car c'est véritablement, à nos yeux, la base du principe républicain. Le projet de loi comporte des dispositions très diverses. En effet, près de 40 sujets différents y sont abordés. En raison de l'urgence, le Gouvernement a demandé à être largement habilité à légiférer par ordonnances. L'Assemblée nationale puis notre commission des lois ont fortement contribué à réduire le nombre d'habilitations, passé de 24 à 10. Nous le saluons.

depuis le début de la crise. En effet, cinq lois ont été votées depuis la fin du mois de mars. Aujourd'hui, l'heure est à la relance. Nous devons tous être mobilisés pour favoriser un retour à la normalité progressive et continue dans notre pays, tout en gardant à l'esprit que nous devrons apprendre à vivre ensemble avec le virus.

d'y apporter son regard, son expérience et, donc, de l'améliorer. La crise sans précédent que nous avons traversée justifie naturellement l'urgence et la rapidité d'examen des différents textes auxquels le groupe Union Centriste a toujours apporté un appui constructif et bienveillant, car notre pays avait besoin de mesures urgentes, qu'elles soient sanitaires, économiques ou sociales. Avec deux lois, une organique et une ordinaire, une loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire et deux lois de finances rectificatives, le Parlement s'est largement mobilisé, même dans des conditions matérielles difficiles. Le Gouvernement, afin de pouvoir agir vite, devait légitimement bénéficier du soutien préalable des législateurs que nous sommes, mais sous l'oeil des parlementaires soucieux du contrôle de l'action gouvernementale que nous ne sommes pas moins. pas moins. Si l'état d'urgence sanitaire est toujours déclaré, nous sommes arrivés aujourd'hui dans une temporalité différente : après la période de confinement qui a nécessité de légiférer rapidement, et donc le plus souvent par ordonnances, nous sommes désormais dans une période de déconfinement progressif, qui doit être celle non pas du maintien de l'état d'exception, mais de la préparation du retour à l'état ordinaire, habituel, pour toute prise de décision démocratique. Ainsi, le recours massif aux ordonnances, tel qu'il était prévu par le projet de loi initial, ne se justifie plus, comme l'a d'ailleurs signifié le Conseil d'État. Ce positionnement a d'abord été repris par nos collègues députés, puis par notre commission des lois. Sous l'impulsion des parlementaires, ce sont entre trois et quatre fois moins d'habilitations à légiférer par ordonnances qui figurent aujourd'hui dans le texte. Les 10 habilitations restantes s'ajoutent d'ailleurs aux 57 ordonnances déjà prises en application de la loi d'urgence du 23 mars dernier. Au passage, il est illusoire d'imaginer que ces dernières seront ratifiées par le Parlement. C'est regrettable, car une habilitation n'a de sens que s'il y a contrôle de son utilisation par la ratification. C'est aussi dommageable à la qualité de la norme,

La notion d'urgence doit donc être prise avec gravité et j'invite chacun d'entre nous à l'utiliser avec parcimonie. J'aimerais, à ce stade, saluer le travail d'analyse et de proposition de nos trois rapporteurs, respectivement de la commission des lois, de la commission des affaires sociales et de la commission des finances, qui ont travaillé avec des objectifs communs que nous partageons

C'est entre ces trois qualificatifs qu'il a fallu choisir pour enrichir et resserrer le texte. Il nous faut néanmoins envisager les dispositions proposées à l'aune d'un double impératif : répondre à la crise par des mesures dont la plupart prolongent des décisions déjà prises et anticiper certaines décisions nécessaires à l'action.

Face à un risque de récession inédite, il est essentiel de relancer notre pays, aujourd'hui à l'arrêt. Les enjeux sont d'importance : il s'agit d'assurer la continuité des services publics et l'organisation des pouvoirs régaliens, de réamorcer la pompe en relançant notre économie tout en évitant que les difficultés des entreprises ne se traduisent par un chômage de masse et par un accroissement des difficultés de nos concitoyens. C'est un enjeu immense. Nombre de mesures proposées nous paraissent nécessaires, qu'elles touchent à la prorogation de divers mandats en dehors du champ politique, à la continuité des missions dans lesquelles nos forces armées sont engagées ou encore à diverses mesures sectorielles touchant, par exemple, aux domaines de la recherche ou du sport. Ce Ce projet de loi répond aussi à un souci de protection des salariés. Je pense notamment aux mesures qui favorisent la reprise de l'activité des entreprises tout en offrant un cadre plus sécurisant aux salariés. En revanche, certaines mesures, comme celles qui sont contenues à l'article 3 et prévoient une mutualisation de la trésorerie de nombreux acteurs publics au sein du Trésor, nous paraissent manquer de préparation et de précision. mutualisation peuvent être entendus, mais il faut travailler à un meilleur encadrement et à une meilleure définition de son périmètre si vous souhaitez la rendre acceptable. En effet, elle pourrait priver plusieurs organismes publics, ainsi que les collectivités territoriales, de ressources induites en rigidifiant leurs mouvements et besoins de trésorerie au seul profit de l'État. Nous devons pouvoir mesurer précisément son impact. Le rapporteur général et de nombreux groupes ont ainsi souhaité sa suppression dès le stade de la commission. Il faut la maintenir. À titre plus personnel, je me réjouis, avec Catherine Di Folco, ma corapporteure du projet de loi de transformation de la fonction publique, que nous ayons pu faire adopter plusieurs amendements visant notamment l'élargissement, hors état d'urgence sanitaire, de la mise à disposition à titre gratuit des agents territoriaux ou hospitaliers auprès des hôpitaux ou des Ehpad, selon la volonté des employeurs publics, ou encore à la « neutralisation » des effets de l'état d'urgence sur la transformation de CDD en CDI dans les trois versants de la fonction publique.

En outre, le Conseil d'État a constaté que l'étude d'impact se bornait à fournir des indications très parcellaires sur certaines habilitations. Même si nous pouvons comprendre les particularités des circonstances actuelles, nous condamnons cette méthode qui nous oblige à discuter, pêle-mêle, des réservistes de la police, des tickets-restaurant, de la justice pénale, des compétitions sportives ou encore des suites des essais nucléaires dans le Pacifique.

Malgré tout cela, à partir du texte déjà amendé dans le bon sens par l'Assemblée nationale, nos commissions des lois, des affaires sociales et des finances ont réalisé un travail considérable et remarquable. Elles ont équilibré les mesures, réduit les durées d'habilitation et amélioré les rédactions juridiques. Pour ces raisons, nous tenons à remercier nos rapporteurs : Mme Jourda, M. Savary et M. de Montgolfier. Ils ont joué le jeu et ont été suivis par leurs commissions dans cette démarche, fidèles à ce qui a toujours été l'un des principaux soucis du Sénat : enrichir et améliorer la loi. malgré cet effort salutaire, il faut bien reconnaître que nous faisons souvent pour le mieux avec ce que l'on nous donne. Une fois le texte promulgué, on s'interrogera sans doute sur sa lisibilité pour nos concitoyens. Même maintenant, ce projet de loi ne brille ni par sa clarté ni par son intelligibilité. Au-delà de ces questions de forme, qu'en est-il du fond du texte ? Nombre de choses, que je ne pourrais guère résumer ici sans risquer de vous ennuyer par un inventaire à la Prévert, qui ne serait qu'une répétition imparfaite de ce qui a déjà été dit. Je ne m'arrêterai donc que sur quelques points, parmi beaucoup qui auraient pu être soulevés. Parfois, le recours aux ordonnances se justifie indéniablement. C'est la raison pour laquelle nous avons voté de larges habilitations le 23 mars dernier. Mais nous ne pouvons que nous interroger face au dépôt d'un texte qui ne comprenait initialement que des ordonnances, alors que nombre d'entre elles pouvaient aisément être immédiatement inscrites dans la loi. Il ne doit pas y avoir de glissement vers un recours systématique à l'ordonnance- à plus forte raison lorsque la procédure allant de l'habilitation à la ratification finit parfois par être plus longue que la procédure législative ordinaire. C'est donc avec satisfaction que je constate que les habilitations ne sont plus qu'au nombre de 10, complétant un processus entamé à l'Assemblée nationale. Il s'agit non pas d'une simple suppression, mais bien d'un enrichissement, car certaines mesures objectivement abouties ont pu être utilement inscrites « en clair » dans la loi.

La commission des affaires sociales, pour sa part, a inscrit dans la loi les habilitations portant sur le prêt de main-d'oeuvre, sur l'indemnisation du chômage et sur la représentation des salariés des TPE. La commission des lois a néanmoins été plus circonspecte sur certains dispositifs. C'est en particulier le cas de l'extension à trente départements de l'expérimentation des cours criminelles. Mme le rapporteur, ce dispositif fait courir le risque de détourner de son objet cette expérimentation pour en faire un simple outil de gestion du stock d'affaires. Laissons donc de côté cette extension problématique afin de pouvoir, le moment venu, procéder à une évaluation rigoureuse de cette expérimentation en fonction de ses seuls mérites. Enfin, l'article 3 a été supprimé par la commission des finances. Il habilitait le Gouvernement, pour une durée d'un an, à prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine législatif en vue de renforcer la centralisation des fonds détenus par certaines personnes morales sur le compte unique du Trésor. La commission des finances n'avait pu obtenir d'informations précises sur les organismes concernés,

Pour conclure, nous avons donc affaire à un projet de loi assez baroque, qui interroge presque plus par sa forme que par son fond. Néanmoins, nous estimons que le travail effectué par les commissions a permis de le bonifier et de le toiletter suffisamment pour le rendre acceptable. C'est sur cette base que groupe Les Républicains votera ce texte. La parole est à Mme Monique

Je commencerai, bien évidemment, par ce qu'il contient. Nous traversons une crise d'une exceptionnelle gravité, qui impose des mesures tout aussi exceptionnelles. Vous en avez pris certaines, comme le chômage partiel qui a probablement évité des faillites en nombre et leur corollaire, les pertes d'emplois- tout du moins Au fur et à mesure qu'apparaissent les difficultés, vous avez besoin d'adapter les différents dispositifs. Si nous comprenons que vous devez agir dans l'urgence, nous n'admettons pas la mise à mal du travail parlementaire, pas plus que celle du dialogue social. Cette frénésie d'habilitations qui mène, entre autres, à une mise aux enchères moins-disantes du code du travail ne peut durer plus longtemps.

Vous affirmez vouloir protéger les salariés les plus précaires et, dans le même temps, vous gravez dans le marbre la libéralisation du régime des CDD. Vous ouvrez aussi la porte à une modification du fonctionnement des comités sociaux et économiques (CSE) et vous permettez l'utilisation des réserves de certains régimes de retraite à des fins d'aides sociales. Certes,

maintenant à ce que ce projet de loi ne contient pas. Depuis le 11 mai dernier, notre pays revient peu à peu à la vie. Lentement, prudemment, mais- espérons-le -sûrement. Ce retour à la vie, comme il est de mise après un cataclysme, est saisissant de contrastes. Celui que je relève en premier et auquel je ne peux m'empêcher de faire référence, c'est le changement de discours du Président de la République : après avoir fustigé sur le quai d'une gare « ceux qui ne sont rien », rend hommage à ces femmes- fort nombreuses -et à ces hommes qui ont tenu le pays depuis le 15 mars dernier en continuant leur travail. Puissent ceux qui les croisent sans jamais les regarder se le rappeler.

Qu'il s'agisse de ceux qui nous ont maintenus en vie, au sens propre comme au sens figuré, ou de ceux qui, demain, seront menacés de dépression économique, il nous faut tracer des perspectives. Pas des perspectives pour après-demain, ni même pour demain, mais des perspectives immédiates. Or ce projet de loi qui arrive au début du déconfinement ne déconfine pas grand-chose. C'est qu'il vous faut, si vous voulez prendre au mot le Président de la République, détricoter à peu près tout ce que vous avez tricoté depuis trois ans, à savoir votre politique fiscale pour remettre enfin un minimum de justice sociale dans ce pays, à savoir votre vision très élitiste de la société, où seule avait droit de cité la « start-up nation à savoir votre réforme du chômage, qui s'avérait déjà fort injuste et qui s'avérera inique dans les circonstances actuelles si vous n'y mettez fin, à savoir votre discours lénifiant sur l'égalité femmes-hommes, qui ne trouvait aucune concrétisation réelle. En fait, monsieur le ministre, madame la secrétaire d'État, nous n'avons pas besoin d'un acte de contrition télévisé dont nous doutons d'ailleurs terriblement de la sincérité. Nous voulons des mesures propres à remettre au coeur de la société ceux qui la maintiennent au quotidien et ceux qui en sont exclus. Le tout par une réforme fiscale courageuse et après un vrai débat parlementaire.

ce projet de loi est un texte fourre-tout, qui pose de sérieuses questions de principe quant aux droits du Parlement. Comme plusieurs d'entre nous l'ont rappelé, la crise sanitaire ne justifie pas tout. Je concentrerai mon intervention sur l'article 4, qui traite du Brexit et que j'ai examiné avec un intérêt particulier en tant que rapporteur de la loi du 19 janvier 2019, dont cet article est en quelque sorte le « petit frère ». La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, bien qu'elle ne soit pas saisie pour avis, en a débattu par visioconférence la semaine dernière. Il s'agit aujourd'hui d'habiliter le Gouvernement à combler les vides juridiques susceptibles d'apparaître à l'issue des négociations en cours entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, notamment si ces négociations devaient échouer. L'hypothèse d'un n'est pas une simple vue de l'esprit les négociations, cela n'aura échappé à aucun d'entre nous, se passent très mal. Des blocages de fond demeurent sur des sujets cruciaux tels que la pêche ou l'équité des conditions de concurrence. Les tensions demeurent vives sur les sujets théoriquement résolus des contrôles à effectuer en mer d'Irlande, des droits des citoyens et des droits de douane. L'impasse devient évidente, les Britanniques ne souhaitant pas prolonger la période de transition. raison pour laquelle je ne suis pas hostile à une habilitation symétrique de celle que nous avions accordée au Gouvernement l'an dernier. Je vous rappelle, mes chers collègues, que toutes

Nous ne pouvons accepter des habilitations « balai » permettant au Gouvernement de combler d'éventuels oublis, alors que cela fait maintenant presque quatre ans, comme vous l'avez rappelé, madame la secrétaire d'État, que nous sommes prévenus qu'il y aura un Brexit.

envisagé de déposer au nom de notre commission. J'apporte donc mon entier soutien à la nouvelle rédaction de l'article 4 issue des travaux de la commission des lois, en particulier au délai d'habilitation réduit à sept mois. En conclusion, mes chers collègues, la crise sanitaire ne doit pas nous faire perdre de vue le Brexit. Les citoyens doivent s'y préparer. Je voudrais redire ici que les ressortissants britanniques restent tout à fait bienvenus sur notre territoire, contrairement à certaines déclarations entendues de l'autre côté de la Manche, vendredi soir dernier. Il doit en aller de même pour les citoyens français au Royaume-Uni.

même quarantaine aux Anglais qui souhaiteraient venir chez nous. Enfin, mes chers collègues, n'oublions pas que les entreprises aussi doivent se préparer, car les conséquences du Brexit viendront malheureusement

Nous cherchons à négocier avec les Britanniques, pour justement conserver le caractère dual, mais unifié, de la commission intergouvernementale sur la sécurité ferroviaire. L'ordonnance n'interviendrait qu'en dernier recours, c'est-à-dire

politiquement, en tant que Parlement uni derrière le Gouvernement, à indiquer aux Britanniques que nous sommes prêts à négocier douze mois de plus, s'ils souhaitent aller dans cette voie. Nous devons faire preuve d'une grande ouverture, parce que, je le répète, un accord coûte que coûte n'est pas ce que nous cherchons.

raison pour laquelle le Gouvernement, pour ne pas revenir devant vous avec la même disposition dans six mois, vous propose de nous faire confiance pour les quinze prochains mois, sur les quatre sujets dont nous parlons.

Je souhaite appeler votre plus grande attention sur la situation exceptionnelle que connaissent de nombreux acteurs du champ artistique et culturel, notamment les établissements publics de coopération culturelle. Alors qu'il leur avait été assuré, mi-avril, qu'ils pouvaient bénéficier du dispositif d'activité partielle, l'ordonnance du 22 avril 2020 les en exclut. Dès le lendemain et à plusieurs reprises les semaines suivantes, le ministre de la culture déclarait : « Nous sommes en train de faire en sorte que toutes ces mesures soient applicables aux établissements publics à vocation industrielle et commerciale relevant des collectivités territoriales. » Le 5 mai, il précisait qu'ils pourraient « désormais bénéficier des aides de l'État

De plus, sur le fond, ce choix, s'il était confirmé, marquerait une rupture économique majeure pour ces établissements, dont les budgets auront à supporter sur plusieurs années les effets du confinement et leur exclusion des dispositifs du chômage partiel. Si l'État ne venait pas en aide à ces structures, il imposerait également une charge supplémentaire aux collectivités territoriales. Enfin, vous ne pouvez ignorer la portée non seulement économique, mais aussi symbolique d'une telle disposition pour un pays profondément attaché aux activités culturelles. Aussi, dans le prolongement des démarches de la présidente de la commission de la culture, Mme Catherine Morin-Desailly, je tiens à appeler votre bienveillance, au-delà des clivages politiques, sur les amendements n 55 et 263 portés par Sylvie Robert, dont l'adoption permettrait de sécuriser l'emploi artistique Ils sont le reflet du travail de fond des groupes mis en place par la commission de la culture, inquiète face à un vrai risque d'écroulement de pans entiers de la culture dans notre pays. Très bien

que d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur plus d'une trentaine de thématiques. Les sujets étaient aussi divers et variés que les règles ayant trait aux CDD, à la prolongation des mandats des conseillers prud'homaux, à l'organisation de la défense française, ou encore aux prérogatives des fédérations sportives pendant la pandémie. Aucun de ces sujets n'est sans importance et la plupart auraient mérité un projet de loi, afin que le Parlement n'ait pas à se délester en urgence de sa compétence à amender les décisions gouvernementales. Fort heureusement, l'Assemblée nationale et le travail en commission au Sénat ont permis de vider pour moitié cet article de sa substance. Ainsi, plusieurs sujets, notamment la question primordiale des étrangers, sont revenus dans le champ des compétences législatives du Parlement, sans nécessiter le recours à l'article 38 de la Constitution. Nous entendons que le droit français offre à l'exécutif la possibilité de légiférer par ordonnance. comprenez que nous sommes en démocratie et que notre système a été bâti sur la capacité du Parlement à contrôler et corriger si nécessaire l'action gouvernementale. Il n'est pas tolérable de nous faire travailler dans ces conditions, sur des sujets disparates, avec une méthode qui bride le législateur dans son pouvoir d'amendement des projets de loi. Souffrez donc,

Didier Marie et Monique Lubin, s'agissant de cet article 1. Je pense en particulier aux mesures relatives à la justice. Voyez-vous, le jury populaire

Il a été décidé qu'il y aurait une expérimentation dans quelques départements, pour mettre en oeuvre des cours criminelles départementales. L'expérimentation suppose qu'on évalue, au bout d'un certain temps, les conséquences de la mesure.

à vous remercier pour reprendre la formulation de Muriel Jourda, destinée à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances. Je veux à mon tour reconnaître le travail de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui ont considérablement réduit le nombre et le périmètre des habilitations.

aussi éloignés et importants que : le fait d'assurer le maintien des compétences et des moyens humains nécessaires à la continuité de l'exercice des missions militaires et de service public ou à la poursuite de l'activité économique

notamment aux caractéristiques des entreprises en fonction de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, de leur secteur d'activité ou des catégories de salariés concernés,

qui s'exonèrent totalement du contrôle du Parlement. L'état d'urgence ne peut justifier de confiner la démocratie. Or le recours étendu et quasi illimité aux ordonnances revient à donner un blanc-seing à un pouvoir qui, déjà, concentre de nombreuses

n'apporte aucune réponse aux conséquences réelles et profondes de la crise sociale, économique et de santé liée au Covid-19.

Ce texte tend à habiliter le Gouvernement à légiférer seul, car nous sommes en état d'urgence. Vous avez voulu prolonger cet état d'urgence jusqu'au 10 juillet inclus ; ce n'était pas mon choix. Ayez la cohérence de n'accorder cette habilitation exceptionnelle que jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire. Je m'étonne que le fait de bafouer ainsi le Parlement ne fasse pas plus bondir les démocrates que vous prétendez être, mes chers collègues On ne légifère pas sans le Parlement. La Macronie a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, et je comprends qu'elle demande une immunité plus longue que prévu. Mais on ne fait pas la loi sans le peuple, ses représentants et les territoires. Pas de restriction de liberté pour la démocratie représentative. Ici, dans cette Haute Assemblée, nous représentons les régions, les départements, les EPCI, plus simplement les collectivités territoriales, les communes, leurs habitants, leurs élus et leurs agents. Dans le mot « collectivités », on entend bien commun, intérêt général, proximité et communauté. Dans le mot « territoriales », on entend terroir, terre, identité, attachement et racines. Entendez-vous et comprenez-vous encore ces deux mots, mes chers collègues ? C'est tout l'inverse de l'individualisme et du progressisme de la « start-up nation ». On comprend dès lors pourquoi ce gouvernement en marche perpétuelle et déraciné cherche à se soustraire au contrôle du Parlement pour plusieurs mois. J'aurais aimé que le Gouvernement, qui nous demande notre aval pour légiférer à tout-va, ait été aussi exemplaire que nos maires ont fait un travail formidable de proximité et d'efficacité, agissant avec un engagement total. Nous sommes ici leurs représentants. Ce sont eux qui sont bafoués par ce programme fourre-tout. La confiance, cela ne se décrète pas, cela se gagne. Moi-même, comme des milliers de maires et des millions de Français, je n'ai pas confiance dans ce gouvernement en sursis. Si vous ne votez pas cet amendement, vous laissez se créer un dangereux précédent pour notre droit. Vous validez un glissement du droit d'exception vers le droit commun. Le monde d'après sera ce que nous en ferons. Là encore, vous serez tenus responsables : ne devenez pas des coupables volontaires Ne dévoyez pas notre démocratie, ne cédez pas vos droits et, surtout, vos devoirs de parlementaires, ne laissez pas le pouvoir jacobin prendre les rênes seul, en écartant le peuple et ses représentants.

à l'exception des dispositions concernant les règles d'activité partielle, pour lesquelles nous donnerions au Gouvernement un délai pour légiférer par ordonnances de six mois, ce qui lui laisserait le temps d'évaluer la situation économique et d'adapter les dispositions. L'amendement

les professionnels, en première ou seconde ligne, mais aussi de tous les bénévoles qui ont continué à faire vivre la solidarité. Les associations ont pu maintenir leurs activités et redoubler d'efforts, malgré des difficultés importantes d'un point de vue logistique, mais aussi économique. À ce titre, je veux rappeler la situation alarmante d'Emmaüs, qui a dû faire appel aux dons pour la première fois depuis sa création. J'espère qu'il y aura une fin heureuse et un engagement massif de l'État. Parallèlement, plus de 260 000 personnes se sont inscrites sur la plateforme jeveuxaider.gouv.fr, intégrant de fait la réserve civique. Malheureusement, cet engagement exemplaire est aujourd'hui en train d'être totalement dénaturé. On le sait, un certain nombre d'entreprises ayant une mission de service public ne pourront pas, dans les semaines qui viennent, reprendre leur pleine activité. L'exposé des motifs du projet de loi évoque notamment La Poste, qui fonctionne à flux tendu depuis des années. Ainsi, l'absence d'un certain nombre de salariés pour des raisons de santé ou de garde d'enfants conduit l'entreprise à de grandes difficultés pour remplir sa mission de service public. La seule solution qu'a trouvée le Gouvernement, c'est de recourir à la réserve civique.

d'autant, faut-il le rappeler ici, que ce dumping social est déjà partiellement à l'oeuvre, avec l'ouverture toujours plus grande des structures d'accueil du service civique, à tel point que l'Agence du service civique elle-même s'inquiète de la recrudescence des emplois déguisés au sein du dispositif. du côté des bénévoles, ils se sont inscrits sur la plateforme et se sont engagés dans la réserve pour faire fonctionner la solidarité et venir en aide aux personnes dans le besoin. Il ne s'agissait pas pour eux de faire fonctionner des entreprises en remplaçant des salariés Les limitations apportées par la rapporteure en commission sont un premier pas, mais nous semblent encore insuffisantes pour régler vraiment le problème. Si on reprend l'exemple de La Poste, les réservistes pourraient se retrouver en position de distribuer le courrier ou la presse ou de tenir les guichets de La Banque postale. Une telle situation pose question, surtout quand on se rappelle la vocation

une bonne partie des secteurs du tourisme, de la culture, du sport ne peuvent pas reprendre leur activité. Il y aura certainement des évolutions dans les jours et les semaines qui viennent, en fonction de la situation sanitaire, mais il est très important pour nous de pouvoir, à compter du 1 juin,

Tout le monde ici est évidemment favorable à une reprise de l'activité : tout le monde souhaite que notre pays redémarre le plus vite possible. Mais nous savons, les uns et les autres, qu'un certain nombre de pans de l'activité resteront malheureusement

l'activité redémarre mais reste encore insuffisante, d'autres salariés ne bénéficient plus de ce dispositif. Je voudrais que vous répondiez à ces préoccupations de telle sorte que nous puissions voter en conscience, considérant

Monsieur le sénateur, pour éclairer complètement notre discussion, je vais être un peu plus précise sur les modalités, les secteurs, les catégories de

nous diminuions la prise en charge dès maintenant : les hôtels, les cafés, les restaurants, les entreprises qui en dépendent, le secteur touristique, l'activité culturelle, l'événementiel, les festivals, les grands événements sportifs seraient

j'en ai bien conscience. Simplement, il faut bien faire attention aux effets pervers quand on prend une mesure économique, notamment quand on prend une mesure que je qualifie volontiers de mise en salariat de la fonction publique de l'ensemble de l'économie française. Il y a là un vrai sujet.

n° 100 rectifié. L'habilitation dont il s'agit tend à autoriser le Gouvernement à apporter des adaptations pour ajuster les dispositions relatives à l'activité partielle, dans le prolongement de l'article 11 de la loi d'urgence du 23 mars dernier. Ainsi, on pourra prévoir la différenciation du dispositif d'activité partielle en fonction des secteurs d'activité pour préserver ceux qui souffrent le plus des effets de la crise sanitaire, comme l'hôtellerie et la restauration.

C'est le cas des fournisseurs ou prestataires de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, qui représentent un certain nombre de TPE et de PME réparties sur l'ensemble de notre territoire. Cet amendement vise à accorder une attention particulière à ces secteurs.

c'est bien beau de dire que l'on va s'intéresser à toutes les filières, dans une logique intégrée. Mais il faut aussi s'intéresser à tous les acteurs des filières ! Je le dis très solennellement. Aujourd'hui, le Président de la République a cru bon

Cet amendement vise à élargir l'applicabilité de l'activité partielle à certains employeurs publics. Or il ne semble pas opportun de prévoir une extension de l'activité partielle dans le cadre d'une habilitation destinée, au contraire, à organiser la sortie progressive

une activité dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. Le Gouvernement considère que cette condition est légitime pour apprécier la prise en charge au titre de l'activité partielle des salariés de droit privé de ces établissements, dans la mesure où ceux-ci bénéficient par ailleurs d'une prise en charge de l'État les subventions d'équilibre ils ne sont donc pas aussi menacés que les autres entreprises commerciales par les difficultés économiques actuelles. Le critère de la part majoritaire des ressources permet de cibler les établissements dont le modèle économique est le plus fortement détérioré. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

de la fin de l'année 2020. En effet, alors que, dans certains secteurs d'activité, les entreprises seront durablement affectées par la crise, le dispositif actuel d'activité partielle, prévu pour répondre à une situation d'urgence, n'a pas été conçu pour un tel accompagnement. Quel est l'avis de la commission

qui permettrait d'accompagner les entreprises subissant une baisse durable d'activité pendant une période plus longue que la simple crise sanitaire, en contrepartie d'engagements, notamment en matière de maintien dans l'emploi, bien au-delà même de 2020. Ce dispositif peut paraître intéressant, mais admettez que la rédaction de l'habilitation est bien vague- trop vague.

Pourquoi devrions-nous voter aujourd'hui une mesure qui s'appliquera dans plus de six mois, dans une configuration économique que nous ne pouvons absolument pas apprécier, tant nous

Or ces questions de droit du travail relèvent non pas de la compétence des fédérations, mais bel et bien de la loi et des dispositions spécifiques au code du sport, ainsi que du dialogue social. Le Gouvernement propose simplement de corriger cette coquille, pour retrouver le sens initial de l'habilitation sur les contrats des sportifs. Cette des sportifs. Cette disposition permettra d'adapter le régime, en particulier la durée des contrats des sportifs et entraîneurs des clubs français, afin de tenir compte des conséquences de l'arrêt des championnats nationaux et de la poursuite d'autres championnats, notamment

Pour répondre à la crise, le Gouvernement prévoit que les accords d'entreprise pourront déterminer le nombre de renouvellements de contrats à durée déterminée. Le nombre de renouvellements possibles pour un CDD, le délai de carence entre deux contrats courts et les cas dans lesquels ce délai de carence n'est pas applicable pourraient désormais être fixés par accords d'entreprise- des assouplissements issus d'un amendement gouvernemental. Les ordonnances Macron de 2017 avaient déjà assoupli le droit en la matière, mais la branche professionnelle restait le verrou. Aujourd'hui, un accord de branche pour déroger au droit du travail, qui prévoit qu'on ne peut renouveler un CDD plus de deux fois. Ce détricotage supplémentaire du code du travail dégrade la qualité de l'emploi et entraînera une précarisation accrue. En favorisant les contrats précaires au détriment des contrats à durée indéterminée, le Gouvernement prétend relancer l'économie. En réalité, il va précariser davantage notre société, d'autant que les mesures présentées comme provisoires deviennent bien souvent permanentes- permanentes- l'excuse a déjà servi par le passé ... Nous sommes particulièrement inquiets d'une disposition qui aggrave les reculs d'une loi que nous avions combattue, la loi El Khomri. L'assouplissement des règles relatives aux CDD et à l'intérim s'est toujours accompagné d'une précarisation des conditions d'emploi pour les travailleurs concernés, concernés, sans effet notable en termes de relance économique. L'argument de la nécessité de s'adapter à la crise est d'autant plus fallacieux que les règles sont déjà largement flexibles et que les employeurs peuvent y recourir facilement

et des représentants des salariés actionnaires dans les organes de gouvernance. Afin d'assurer la continuité de cette représentation essentielle, le présent amendement tend à proroger les mandats des représentants qui ont expiré sans pouvoir être renouvelés ou remplacés en raison du contexte sanitaire. En outre, pour offrir une souplesse aux entreprises confrontées aux difficultés matérielles d'organisation de ces élections, l'amendement vise à aménager la date limite d'entrée en fonction des représentants qui devront être désignés à la suite du renforcement des obligations de représentation des salariés et des salariés actionnaires par la loi Pacte.

au 31 décembre 2020 ou à trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, si cette date était postérieure au 30 septembre

: le recours facilité aux contrats précaires ne permettra pas d'améliorer la situation économique du pays. Au reste, ces mesures s'appliquent déjà depuis des années, sans succès.

l'amendement n° 5 rectifié . Dans la période de crise actuelle, le maintien des salariés en parcours d'insertion revêt un intérêt particulier pour éviter une exclusion durable du monde du travail en conservant un lien avec l'employeur, qui peut poursuivre son action d'accompagnement et de formation dans l'attente de la reprise d'activité. Le Gouvernement a souhaité faire bénéficier l'ensemble des salariés de la mesure renforcée d'activité partielle afin de préserver l'emploi face à cette crise. Pour autant, en raison de particularités juridiques, les associations intermédiaires et les entreprises de travail temporaire d'insertion voient leur accès à cette mesure de soutien remis en cause en raison d'une insécurité juridique liée à la nature de leurs contrats d'insertion. Le présent amendement, proposé par Mme Delattre, vise donc à adapter l'accès à l'activité partielle à la particularité des contrats à durée déterminée d'usage d'insertion.

que l'insertion par l'activité économique puisse bénéficier du chômage partiel. Cela nous semble une bonne chose compte tenu de la crise actuelle. La parole

compte tenu de la spécificité de ces structures. Ces amendements sont satisfaits par la pratique actuelle de la DGEFP, qui est précisée dans une simple foire aux questions du ministère du travail. Cependant, on voit mal pourquoi cette pratique ne serait pas sécurisée juridiquement.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Conscient de la particularité du secteur de l'insertion, pour lequel il importe de garantir la continuité des parcours individuels et d'éviter toute rupture de prise en charge, le ministère du travail a très tôt indiqué la possibilité pour les structures d'insertion de renouveler à titre exceptionnel les CDDU arrivés à échéance.

du 25 mars 2020 a ouvert des dérogations dangereuses au droit du travail en matière de congés payés et de jours de repos pour tous les secteurs, ainsi que des dérogations concernant la durée maximale du travail et le repos dominical. Les entreprises n'ont pas attendu pour mettre en place ces dispositifs, y compris les grands groupes qui bénéficient déjà du chômage partiel et des aides financières de l'État. Je pense à Alstom, qui a imposé à ses salariés de poser avant fin avril onze jours de repos, dont cinq jours de congés payés. Ces salariés n'ont pas eu le choix de leurs jours de congé,

Chez BNP Paribas, la direction a imposé unilatéralement la prise de dix jours avant fin mai. Cette décision brutale a été extrêmement mal vécue par les salariés. vécue par les salariés. Certaines entreprises ont également imposé à leurs salariés de réduire ou de déplacer leurs congés d'été. Ainsi, chez PSA, un accord diminue de trois à deux semaines consécutives la durée minimale des congés estivaux. Cette remise en cause brutale des congés d'été est une double sanction pour les salariés, qu'ils aient été confinés aient continué de travailler sans beaucoup de protection. Par l'ordonnance de mars 2020, une brèche supplémentaire a été ouverte au socle des droits sociaux de notre pays. Le risque est de voir cette brèche maintenue au-delà du 31 décembre 2020. Pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons

? Ces trois amendements tendent à revenir sur les mesures d'urgence en matière de congés et de temps de travail. L'amendement n° vise à abroger l'ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, qui a été prise sur le fondement de la loi d'urgence du 23 mars. Les mesures de cette ordonnance relatives à l'adaptation des règles de prise des congés payés ont donné lieu à de nombreux accords collectifs sans susciter d'opposition majeure. Elles permettent aux entreprises de s'organiser en vue de la reprise de l'activité économique. Supprimer ces mesures aujourd'hui poserait un problème de sécurité juridique. Par ailleurs, les dérogations aux règles de durée de travail n'ont à ce jour donné lieu à aucun décret sectoriel.

et 205 rectifié visent à supprimer des habilitations sur le fondement desquelles a été prise cette ordonnance pour permettre aux employeurs de déroger respectivement aux règles de prise de congés payés et de jours de repos et aux règles d'ordre public

cas, permet aux entreprises de faire face aux difficultés économiques liées à la pandémie de Covid-19 et participe ainsi de l'aide indispensable au tissu économique et au maintien de l'emploi des salariés en entreprise.

de ce dispositif, comme l'a rappelé votre rapporteur pour avis. De nombreux accords de branches et d'entreprise ont déjà été signés. Le dispositif est donc jugé pertinent et adapté par les forces économiques et sociales sur le terrain. J'émets donc un avis défavorable sur l'amendement n°

la mise en oeuvre de deux mécanismes visant à compléter les revenus des salariés dans le cadre d'un placement en activité partielle. Le premier mécanisme permet à l'employeur d'organiser une solidarité entre les salariés de l'entreprise de façon à monétiser les jours de repos et les jours de congés payés de ceux qui n'ont pas subi de perte de rémunération vers ceux qui qui ont vu leur rémunération diminuer du fait de leur placement en activité partielle. Le second mécanisme, qui repose sur le volontariat des salariés, vise à permettre aux salariés qui ont subi une baisse de leur rémunération du fait de leur placement en activité partielle de compléter leurs revenus par la monétisation de jours de repos ou de jours de congés payés. Dans les deux cas, seuls les jours de repos conventionnels et les jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine peuvent faire l'objet d'une monétisation. sociales ? L'idée de monétiser des jours de congé ou des jours de repos non pris pour maintenir la rémunération des salariés placés en activité partielle semble dans le contexte actuel très positive.

trouver à s'appliquer dans de nombreuses entreprises dans lesquelles l'indemnisation de l'activité partielle est variable selon les catégories de salariés. Le dispositif de fonds de solidarité pourrait être imposé par l'employeur, mais il serait conditionné à la conclusion d'un accord d'entreprise, ce qui constitue une garantie qui nous paraît suffisante. Le droit actuel a déjà permis à de nombreuses entreprises de conclure des accords innovants pour faire face aux conséquences de l'épidémie. Cet amendement peut leur permettre d'aller plus loin. L'avis est donc favorable.

Le Gouvernement est favorable aux deux mesures proposées, qui permettent l'une et l'autre le maintien de la rémunération des salariés en activité partielle. La mise en place d'un fonds de solidarité par accord collectif permettra aux partenaires permettra aux partenaires sociaux de déterminer les conditions de mise en oeuvre du mécanisme les mieux adaptées à l'entreprise. La monétisation des jours de repos et exceptionnellement de la cinquième semaine de congés payés, dans le respect des engagements européens, qui prévoient que les quatre premières semaines de congés payés sont prises sous forme de repos,

Toutefois, cette décision est désormais lourde de conséquences à long terme et risque d'affaiblir un peu plus la place du sport, particulièrement du football français sur la scène européenne et de le rendre ainsi plus vulnérable face à la concurrence des grands championnats voisins. Les enjeux sont multiples, notamment économiques. La perte est estimée à plus de 700 millions d'euros. Cette décision provoque donc une certaine incompréhension, d'autant plus que plusieurs pays européens ont fait des choix radicalement différents. Un sportif différents. Un sportif de haut niveau a besoin de cinq à six semaines d'entraînement intensif pour être en forme physiquement. Par ailleurs, pour éviter une chute trop brutale du nombre de licenciés, il faut travailler sur des protocoles de reprise par discipline. discipline. Permettre à nos jeunes de pratiquer leur activité sportive favorite nous évitera d'assister à des organisations sauvages regroupant illégalement des centaines de personnes comme on a pu le voir ce week-end. Pour en revenir à l'économie du sport, si le plan Tourisme dévoilé par le Premier ministre le 14 mai dernier comprend un certain nombre de mesures utiles et bienvenues à la préservation de la filière sport, celles-ci doivent cependant être renforcées pour éviter qu'un trop grand nombre de clubs ne soient menacés. Madame la ministre, merci de nous apporter une réponse claire pour rassurer tous les sportifs, ... Il faut conclure ! ... les nombreux dirigeants et bénévoles des 360 000 clubs, les 112 000 entreprises du sport et leurs 448 000 salariés.

rédaction a été élaborée en concertation avec les acteurs du sport et qu'elle apporte des précisions supplémentaires par rapport à la proposition que vous faites, puisqu'elle intègre une modification des règles spécifiques aux manifestations de sport amateur et des règles sur les conditions administratives et financières des clubs.

1 B pour le secteur du sport. Au regard de la situation exceptionnelle que nous vivons, nos fédérations et nos ligues ont été contraintes de mettre un terme définitif à leurs compétitions sportives pour la saison 2019-2020. Environ un tiers des rencontres et des matches qui restaient encore à disputer Au niveau amateur comme professionnel, les ligues et les fédérations ont dû prendre des décisions sur la fin des championnats et sur les dates ou sur les conditions d'accession ou de relégation entre deux divisions, avec des conséquences sportives qui n'ont évidemment pas satisfait tous les clubs,

Je souhaite également lever une ambiguïté, soulevée lors du débat à l'Assemblée nationale, concernant les décisions que les fédérations et les ligues professionnelles pourraient prendre au titre de la saison 2020-2021 et jusqu'au 31 décembre 2020. Le texte prévoit que leurs instances dirigeantes auront la possibilité de tirer les conséquences d'éventuels forfaits des clubs dans les poules qui seront constituées en début de saison, de tels forfaits pouvant impacter les règles de repêchage ou le format des championnats. En effet, à ce stade, plusieurs clubs, notamment de niveau intermédiaire, sont encore dans l'incertitude quant aux conditions dans lesquelles ils pourront débuter la saison prochaine. Nous souhaitons laisser

Quelles sont les raisons qui ont poussé le Gouvernement à faire le choix d'arrêter totalement les compétitions professionnelles ? Pourquoi avoir pris une décision aussi rapide, sans aucun échange avec les acteurs concernés ?

Nous vous avons interrogée en ce sens, madame la ministre, mais de nombreuses questions restent en suspens. Le sens de mon amendement est clair : il vise à donner la possibilité d'envisager une reprise de la saison actuelle, sous réserve bien sûr d'un avis du comité de scientifiques ainsi que d'un protocole sanitaire adapté.

de loi. Si, dans quelque temps, en pleine crise économique et sociale, on nous demande de voter des aides de l'État- c'est-à-dire des contribuables -d'un montant de plusieurs centaines de millions d'euros pour sauver le foot français, je veux être sûr et certain que les bonnes décisions auront été prises au bon moment et par les bonnes personnes.

mais pas au niveau français. C'est un peu surprenant. Ensuite, il n'est pas question que nous nous immiscions dans les décisions des ligues et des fédérations.

madame la ministre, jusqu'à atteindre un résultat déplorable pour notre pays sur le plan sportif. Vous en porterez la responsabilité devant les 17 millions de nos concitoyens licenciés, les 17 millions de Français qui pratiquent un sport sans être licenciés, tous ceux qui aiment le sport et qui aiment regarder le sport français

Certaines ligues ou fédérations ont d'ores et déjà annoncé des dates de reprise pour leurs championnats. C'est une bonne chose, mais sur quels fondements ces annonces reposent-elles ? Je n'ai pas entendu parler d'un quelconque avis scientifique sur le sujet, ce qui, au regard de l'enjeu, me semble très important.

au regard des enjeux sanitaires et économiques, il me semble déterminant que les décisions du Gouvernement en la matière fassent l'objet d'une véritable analyse scientifique et d'une véritable concertation avec les acteurs concernés.

habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour répondre au caractère urgent d'une crise sanitaire exceptionnelle. Le reste, c'est du hors sujet ou, en tout cas, il devrait en être ainsi. Les étrangers ayant une carte de séjour portant la mention « étudiant » continuent à être assistés par les aides de notre pays, qui sait se montrer si généreux avec les autres, sacrifiant trop souvent les siens. Il est de notoriété publique que la précarité étudiante s'aggrave de jour en jour, et pas seulement pour les étudiants étrangers. Cependant, quand le marché entend le mot « étudiant » ou encore le mot « étranger », il entend « main-d'oeuvre à bas coût Ainsi, vous voudriez permettre aux étudiants étrangers d'exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % du temps de travail annuel : il s'agit véritablement d'une filière déguisée pour le travail saisonnier étranger et une concurrence de l'intérieur imposée à nos compatriotes. Cela va peut-être vous surprendre,

Je demande donc la suppression de cet article.

portant la mention « étudiant » est autorisé à travailler à 60 % de la durée de travail annuelle. Par cet article 1 , le Gouvernement nous propose d'augmenter cette durée de travail à 80 % de manière dérogatoire jusqu'à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur. Nous ne pouvons, hélas, nier la situation de nombre d'étudiants étrangers. Leur quotidien est précaire et leurs ressources particulièrement faibles. Ce dispositif est à double tranchant : certes, il pourrait constituer un complément de revenus non négligeable pour les étudiants étrangers, mais il est également représentatif de la manière dont le Gouvernement aborde la question des migrants sur son territoire. Pour l'exécutif, l'étranger ne saurait bénéficier de véritables droits. Ceux-ci devraient donc être dérogatoires, partiels, temporaires, conditionnés à une conjoncture spécifique et utiles à l'économie française. Nous estimons au contraire que l'État devrait être garant de toutes les personnes touchées par la précarité. Il est donc de son devoir de sécuriser les droits des étudiants étrangers et de ne pas les conditionner à l'urgence sanitaire. Nous souhaitons, par cet amendement, faire en sorte que le dispositif ici présenté n'ait pas une application limitée dans le temps, mais soit inscrit de manière pérenne et durable dans le Ceseda.

! Au contraire, soutenons les agriculteurs qui emploient des Français, grâce à des primes ou l'incitation fiscale ! Les Français sont courageux, ils sont travailleurs. Arrêtez de les faire passer pour des fainéants, comme l'a si bien et si scandaleusement exprimé Emmanuel Macron Encourager l'immigration, c'est encourager le regroupement familial et, donc, laisser s'installer chez nous des gens qui vont profiter de notre modèle social. Nous le savons, celui-ci est le plus généreux et, en conséquence, le plus suicidaire du monde. Où sont les bonnes résolutions du confinement ? Au plus fort de la tempête, quand le Gouvernement sentait la peur d'être submergé par la vague, nous étions en guerre. en guise de testament, venaient se confesser chacun leur tour. On entendait alors parler de patriotisme, de solidarité nationale, de souveraineté nationale. La frontière devenait bienveillante ; la communauté nationale, une réalité. L'Union européenne a prouvé qu'elle était une chimère, inutile et inefficace, mais, l'été arrivant, la vision du front s'éloignant, vous voilà à chercher de la main-d'oeuvre saisonnière au-delà de nos frontières L'article que nous examinons prévoit de prolonger de six à neuf mois la durée de séjour et de travail des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier ».

Bref, toujours plus de main-d'oeuvre à bas coût, et on ne se donne pas les moyens de remettre en activité des travailleurs français ! Pour vous, ils sont trop chers, trop exigeants et trop protégés par le droit du travail. que voulez-vous, nos compatriotes souhaitent une rémunération à la hauteur de l'effort fourni. C'est sans doute trop demander pour un certain patronat « en marche » et un système fiscal français devenu le plus socialiste et, donc, le plus confiscatoire du monde. Ou quand on unit le pire de la droite et le pire de la gauche La précarité de nombreux Français, accentuée par la crise sanitaire, économique et sociale actuelle, exige que le principe de priorité nationale soit de mise pour le travail saisonnier et que tous les moyens soient employés pour permettre aux travailleurs français en difficulté d'obtenir un emploi. La situation actuelle exige une main-d'oeuvre